l'avion. Cette absence totale de contribution sur le carburant des avions est une incongruité en termes d'écologie,

le législateur d'instaurer un régime normal pour les vols intérieurs. En effet, l'avion est aujourd'hui le mode de transport qui émet le plus de C02 par passager transporté.

Les passagers des vols intérieurs métropolitains, hors liaisons soumises aux obligations de service public, appartiennent majoritairement aux catégories socio-professionnelles élevées. Ils sont donc peu sensibles au fameux « signal prix » qui motive en général toute taxation à visée à visée écologique. La mesure n'aura par conséquent que très peu d'incidence sur la fréquentation des lignes et, partant, sur l'emploi. Il s'agit de rétablir une fiscalité plus conforme aux objectifs de lutte contre le changement climatique, réaffirmés entre autres lors de la COP21 il y a trois ans. Il s'agit aussi, indirectement,

de 50 % d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2005 l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'un engagement volontaire de cette industrie ;

les machines-outils, les engins de chantier, les engins de carrière et un certain nombre d'autres véhicules fonctionnant au gazole non routier ne vont pas passer du jour au lendemain à une autre forme d'énergie.

Par ailleurs, il tire également les conséquences de la création du B10 pour ce qui relève de la possibilité prévue pour les conseils régionaux, l'Assemblée de Corse et le Syndicat des transports d'Île-de-France de majorer une fraction du tarif de TICPE. Pour des raisons techniques, cette mesure de régionalisation pourrait s'appliquer à compter du 1 juillet 2019. L'amendement

et apportera une réponse appropriée à la crise actuelle liée à la hausse de la fiscalité sur les carburants. Il s'agit d'une simple disposition de cohérence par rapport à un dispositif fiscal existant

Autorisé depuis mars 2018, le B100 est un carburant contenant jusqu'à 100 % de carburant renouvelable produit à partir de colza. Destiné uniquement aux flottes captives, il constitue une alternative entièrement substituable au gazole et une réponse immédiate aux efforts du secteur des transports routiers

dans les carburants pouvant faire l'objet d'un remboursement pour les exploitants de taxi, les transporteurs routiers de marchandise, les exploitants de transports en commun de voyageurs, de sorte que ce carburant bénéficie du même mécanisme de remboursement d'une fraction de TICPE que le carburant B7.

grandes consommatrices d'énergie bénéficient d'un taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la TICGN. Toutefois, la rédaction de la législation actuelle prive du bénéfice de ce taux réduit certaines entreprises de secteurs d'activité de niche, comme celle des légumes déshydratés, car elles ne correspondent pas aux critères. La difficulté, c'est qu'il s'agit d'un secteur très étroit.

particulièrement en milieu rural, et fait travailler plus de 75 agriculteurs locaux payait, en 2014, 95 000 euros de TICGN et, en 2017, 395 000 euros. En 2018, elle acquittera, 567 000 euros et 1,1 million d'euros en 2022. Les chiffres sont assez parlants. Du fait de la progressivité de la TICGN, ces entreprises ont des seuils de rentabilité très faibles. Il est essentiel de prendre en compte l'importance d'une mesure spécifique pour un secteur très fragilisé, qui a été omis de toutes les discussions par le passé. La fédération professionnelle s'est rapprochée de la Commission européenne pour intégrer son secteur à la liste révisée qui s'appliquera pour la période 2021 à 2030. Nous avons saisi, avec notre collègue Jean Bizet, les ministres de Bercy, en appelant leur attention sur les difficultés de cette filière. Il nous a été répondu qu'ils y étaient très attentifs. Nous avons également saisi le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et l'énergie, M. Miguel Arias Canete, dans la perspective de la révision. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'en est ouvert au ministre Gérald Darmanin en juin dernier. Le législateur doit s'emparer de ce sujet qui concerne le maintien d'activités liées à la diversification de la production agricole, donc exercées en zone rurale, et éviter ainsi que ne se retrouvent dans nos assiettes que des légumes déshydratés d'importation, provenant de Chine, d'Inde, des États-Unis et d'Égypte, avec tous les risques liés à la présence de pesticides en plus, si j'ose dire.

souvent de l'absence de tels services. Sans négliger les autres missions qu'ils effectuent- environ 748 600 interventions -, ces secours impliquent autant de déplacements. Pourtant, dans un contexte de fonctionnement à flux tendus avec des baisses de budgets, les SDIS continuent de payer en totalité le carburant nécessaire à leur intervention, alors que certaines entreprises en sont exonérées ou sont remboursées. Le 6 mars 2018, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics s'est exprimé en défaveur d'une suppression ou d'une exonération en matière de fiscalité sur les carburants. Il ne s'agit pas, aujourd'hui, de revenir sur ces déclarations, mais de proposer un compromis vertueux. un compromis vertueux. La fiscalité sur les carburants est composée pour partie de la TICPE et de la TVA. Le présent amendement a pour objet un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé pour les interventions des véhicules des sapeurs-pompiers. Ce remboursement existe déjà pour les services de transports publics routiers en commun de voyageurs. Les sapeurs-pompiers concourant à l'exécution d'un service public vital, il n'est pas normal qu'ils ne puissent pas en bénéficier aujourd'hui.

les charges qui pèsent sur les SDIS, compte tenu de leur apport fondamental à l'intérêt général et à la solidarité nationale. Le régime d'imposition à la TICPE est toutefois encadré

défendre l'amendement n° I-843. Dans le cadre de leur activité agricole, les exploitants sont fréquemment amenés à sécher leurs productions pour leur permettre d'être aux normes contractuelles et d'assurer une bonne conservation, notamment pour l'exportation.

au remboursement partiel aux entreprises effectuant pour le compte d'exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire la prestation de séchage de grains et de céréales.

Schillinger. Par cet amendement, je propose de renforcer le soutien financier apporté à nos concitoyens, notamment les plus modestes, pour l'achat d'un véhicule propre. Le Gouvernement a déjà mis en place des aides spécifiques. Ainsi, depuis cette année, le montant de la prime à la conversion, basée sur le barème de la vignette Crit'Air, s'élève à 2 500 euros pour une voiture électrique ou à hydrogène, et à 1 000 euros pour les modèles Crit'Air 1 ou 2, dont font notamment partie les véhicules hybrides rechargeables. En cas d'acquisition par un ménage non imposable, la prime est doublée et va jusqu'à 2 000 euros. J'ajoute que, pour les voitures électriques, cette prime à l'acquisition est cumulable avec le bonus écologique, fixé à 6 000 euros en 2018. Ces aides représentent un montant important, mais il faut bien reconnaître qu'en l'état actuel du marché automobile, le prix d'achat des véhicules propres est excessivement plus élevé que celui des véhicules thermiques, de sorte que le passage aux véhicules propres reste hors de portée d'un trop grand nombre de nos concitoyens. Pour accélérer la conversion du parc français, je propose donc d'instituer un dispositif de prêt à taux zéro d'un montant de 7 000 euros, sous conditions de ressources. Ce dispositif sera complémentaire des primes, qui sont souvent versées des mois après l'achat du véhicule. J'ajoute que le décret précisant le mécanisme de prêt à devra veiller à ce que la durée du prêt soit suffisamment longue pour permettre des mensualités de remboursement raisonnables. Cette mesure me semble en cohérence avec notre volonté commune de réussir la transition écologique sans opposer environnement et pouvoir d'achat.

un véhicule électrique consomme plus de CO2 qu'une voiture à moteur thermique.

est 3 500 fois supérieure aux normes tolérées pour l'essence terrestre. L'emploi du gaz naturel liquéfié, le GNL, permet une réduction des émissions de soufre à hauteur de 99 % et une diminution de 20 % des émissions de dioxyde de carbone. Le Gouvernement a fait le choix de soutenir la transition énergétique en faveur du GNL par un dispositif de suramortissement fiscal. L'objet de cet amendement est d'allonger jusqu'au 1 janvier 2025

provoquer un ajustement des choix en matière d'achat de bateaux. Il tient compte de la durée de construction des biens. Il est ouvert aux navires dont le contrat de construction est conclu entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 2021,

conscient de la nécessité d'encourager l'utilisation de carburants alternatifs, le Gouvernement est en train de travailler sur un dispositif de suramortissement pour certains engins non roulants

fait aujourd'hui l'objet d'une non-application de la contribution au service public de l'électricité, la CSPE. Or il apparaît que la législation en vigueur ne permet pas aux situations où l'autoconsommation est réalisée par un mécanisme de tiers payant une non-application de la CSPE, sauf

pour les futurs autoconsommateurs. Le présent amendement vise à simplifier ce mécanisme et à envoyer un signal clair aux entreprises comme aux particuliers,

La parole est à M. Antoine Lefèvre. L'électricité solaire est l'un des atouts de notre territoire pour réussir la transition énergétique. L'une des tendances de fond de la production solaire est la volonté grandissante des citoyens comme des entreprises de pouvoir autoconsommer leur propre production. Cette solution, vertueuse, permet une contribution en nature au verdissement du mix et à la moindre consommation consommation d'électricité issue du réseau. Dans ce cadre, l'autoconsommation individuelle fait l'objet d'une non-application de la contribution au service public de l'électricité et des taxes locales de manière encadrée, au titre de l'article 266 C du code des douanes. Le présent amendement a pour objet d'étendre l'exonération sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité lorsque l'autoconsommation est réalisée en tiers-investissement ou par un ou plusieurs producteurs d'électricité liés entre eux au sein d'une personne morale. Considérant la contribution en nature aux objectifs de transition énergétique et les bénéfices du partage des électrons solaires entre plusieurs consommateurs, permettant ainsi un meilleur taux d'autoconsommation par le foisonnement des usages, il y a lieu d'étendre l'application de l'exonération à l'ensemble des opérations d'autoconsommation collective telles que prévues par le code de l'énergie.

Dans le prolongement des amendements précédents, l'objet de celui-ci est double : favoriser le recours au tiers-investissement dans la filière photovoltaïque et accompagner la transition énergétique dans le secteur industriel. d'étendre le niveau d'exonération de CSPE pour y inclure les installations d'une capacité de production inférieure à cinq mégawatts et non plus uniquement de un mégawatt. Cette mesure permettrait d'encourager le développement des installations d'autoconsommation au sein des sites industriels équipés d'une cogénération tout en réalisant des économies budgétaires significatives. Le présent amendement vise à inclure les situations d'autoconsommation opérées une opération de tiers-investissement dans les cas ouvrant droit à une exonération de CSPE.

Dans certains cas, comme celui des locataires d'habitats collectifs, notamment sociaux, la production d'énergie partagée le réseau public de distribution d'électricité entre plusieurs consommateurs réunis au sein d'une personne morale est la seule manière de produire et de consommer l'électricité solaire

pas répondre à l'objectif d'une meilleure transition vers l'énergie solaire ou les énergies renouvelables. Cette proposition est également incompatible avec le droit européen régissant les taxes pour les motifs que j'ai soulignés tout à l'heure.

le maillage du réseau électrique français, qui constitue un modèle pour beaucoup de pays.

pour recharger un portable, avoir de la lumière et se connecter au monde. La

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

cet amendement permettrait ainsi d'atteindre les objectifs européens de 10 % d'énergies renouvelables en 2020. Enfin, dans le respect des principes de lisibilité, de transparence et de cohérence, le dispositif proposé permettrait d'instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. En effet, le carburant ED95, composé de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, est déjà éligible au mécanisme en cause. En outre, afin de garantir une utilisation exclusive du B100, cet amendement a pour objet d'instaurer des modalités de contrôle qui seront déterminées par les administrations compétentes. À titre d'exemple, les systèmes de contrôle suivants pourront être mis en place, et ce d'autant plus facilement que le B100 est uniquement autorisé pour un usage en flotte captive : l'obligation de recourir à des systèmes de « badging

Par cet amendement, il est proposé d'étendre l'application du dispositif de suramortissement aux véhicules qui utilisent exclusivement du B100. Cet amendement est cohérent avec la stratégie du Gouvernement, le développement du B100 participant pleinement à la transition énergétique. En outre, afin de garantir une utilisation exclusive de ce carburant, il tend à instaurer des modalités de contrôle à déterminer par les administrations compétentes.

qui entrent en zones urbaines et réalisent des kilométrages plus faibles, ce qui rend plus compliqué l'amortissement de véhicules propres plus chers. L'extension jusqu'aux 19 tonnes permet de favoriser la mutualisation des transports et de garantir des gains environnementaux plus importants pour les véhicules desservant les centres-villes. Enfin, le développement des véhicules roulant au gaz naturel pour véhicule est très dynamique pour ce qui concerne les véhicules de plus de 3,5 tonnes. C'est pourquoi il faut concentrer les efforts sur l'ensemble des moyens de transport pour tous les véhicules à deux essieux. deux essieux. L'élargissement de l'application du suramortissement jusqu'aux 19 tonnes permet justement de simplifier la disposition en englobant l'ensemble des véhicules à deux essieux. Une politique cohérente doit prendre en compte le nombre d'essieux, et pas seulement la capacité de transport. Instaurer un seuil à 19 tonnes aurait pour conséquence de créer un dispositif à la fois simple et efficace.

Les exploitants de taxis qui souhaitent acquérir des véhicules électriques bénéficient déjà d'une aide financière accordée par l'État, le bonus écologique. Créer un suramortissement pour les véhicules légers fonctionnant à l'électricité reviendrait à attribuer un double avantage

ayant pour objet d'évaluer les incidences du mécanisme de bonus-malus, dont les flux financiers sont retracés dans le compte d'affectation spéciale « Aide à l'acquisition de véhicules propres », sur la structure des ventes de voitures particulières sur le territoire français et la moyenne des émissions de dioxyde de carbone des véhicules neufs vendus en France. Il s'agit d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement dans le contexte des évolutions successives du barème du malus automobile et du renforcement par le Gouvernement de la prime à la conversion pour les ménages modestes, de même que pour les gros rouleurs. Les données ainsi présentées permettront tout à la fois de fonder et d'éclairer les modifications à venir du malus automobile et des aides à la conversion. L'objet de ce dispositif est donc de nous aider, collectivement, à mieux piloter les dispositions qui ont été récemment mises en place pour accompagner la transition écologique et énergétique s'agissant des motorisations des véhicules.

depuis plusieurs années maintenant, et quel que soit le gouvernement, on a l'habitude de voir des taxes créées sous couvert de transition écologique, dont les recettes sont le plus souvent détournées vers le budget général.

L'article 8 vise à renforcer et à rationaliser la composante « déchets » de la TGAP, afin d'inciter les apporteurs de déchets, publics et privés, à privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d'incinération. À cet effet, il renforce la trajectoire d'augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025, de telle sorte que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets, et il supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d'incinération incompatibles avec cet objectif. Or l'augmentation des tarifs de la TGAP aura nécessairement un impact sur les services publics locaux de gestion des déchets et présente l'inconvénient d'être supportée par les apporteurs de déchets, en particulier les collectivités territoriales et les ménages, qui ne représentent qu'un peu plus de 10 % du total des déchets produits. Elle est en outre particulièrement injuste et précipitée, car la moitié des déchets aujourd'hui éliminés est composée de produits non recyclables, ce qui relève de la responsabilité des metteurs sur le marché, et non des collectivités et des contribuables.

très en amont du projet de loi de finances, lorsqu'il a dévoilé sa feuille de route pour l'économie circulaire. De notre point de vue, la nouvelle trajectoire de la TGAP déchets et la suppression de ces nombreux tarifs réduits sont indispensables pour inverser la hiérarchie des coûts entre les solutions de traitement des déchets. Elle permet aussi, par un signal prix clair, que les flux de déchets soient dirigés de manière prédominante vers le recyclage, plutôt que vers le stockage ou l'incinération.

est à M. Olivier Cadic. Le projet de loi de finances pour 2019 désigne « les matériaux d'isolation ou de construction contenant de l'amiante ». Il est proposé de reprendre la terminologie « déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante », laquelle est employée dans l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Une harmonisation des terminologies permettrait d'assurer une interprétation exacte

Or ces derniers sont produits en grande quantité sur les chantiers de rénovation et doivent être éliminés en installation de stockage de déchets dangereux. Le présent amendement vise donc à étendre la dérogation de TGAP à ces déchets pour lesquels il n'existe pas de filière de recyclage.

Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Morin-Desailly, est très important. En effet, la réforme de la TGAP va à l'encontre d'une politique fiscale incitative et efficace en matière de promotion de l'économie circulaire.

largement à l'effort de recyclage et de valorisation des déchets. J'ajoute que la société française Tree Waste vient de remporter un prix des Nations unies, délivré par la division dirigée par l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy,

dispositifs. La mesure proposée rendrait la valorisation énergétique moins onéreuse que le recyclage. Il nous semble qu'il faut avoir un ordre de préférence : d'abord le recyclage, qui constitue la meilleure pratique,

Je veux simplement rappeler que le rôle de la valorisation énergétique des déchets dans l'économie circulaire a fait l'objet d'un rapport de la Commission européenne, appelant à la poursuite des objectifs du plan d'action de l'Union européenne pour l'économie circulaire adopté en 2015.

1 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour l'État d'ici à 2025. Je rappelle que les recettes de TGAP s'élevaient à 450 millions d'euros en 2017 et devraient donc atteindre 800 millions d'euros en 2025.

la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée

rectifié. Les collectivités n'ont de prise ni sur la conception des produits qui n'ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l'élimination de ces déchets pour lesquels il n'existe aucune alternative.

sur les résidus de déchets non valorisables issus d'installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes. L'objectif est de diminuer le coût des opérations de tri et de recyclage en réduisant le montant de TGAP dû sur les résidus qui ne peuvent pas être valorisés, et qui sont donc envoyés vers des installations de stockage ou d'incinération. Cet abattement ne pourra bénéficier qu'aux installations performantes, dont le volume de résidus est inférieur à un seuil fixé par arrêté. Cet amendement va plus loin que celui du Gouvernement, adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, qui tendait à instaurer un tarif réduit de TGAP sur les seuls résidus de tri à haut pouvoir calorifique traités dans des installations de valorisation énergétique à haut rendement. Une telle mesure est insuffisante, compte tenu de l'absence, dans de nombreux départements, de solution d'incinération à haut rendement, ou de la saturation des capacités de ces incinérateurs, qui conduisent à ce que ces résidus soient orientés vers des installations de stockage. La parole

Cet amendement est le fruit du travail réalisé par les collectivités. Les installations de tri qui sont mises en place

instaurer un abattement de 50 % de TGAP sur les résidus de déchets non valorisables issus d'installations de tri, de recyclage et de valorisation performantes. Il s'agit de réduire le coût des opérations pour les collectivités dont le budget est fortement affecté par la TGAP. amendement va dans le sens de notre proposition de mettre en place une TGAP « amont » qui permettrait de taxer à la source de la production des déchets les metteurs sur le marché, plutôt que les collectivités en bout de chaîne.

qu'à l'heure où le Gouvernement demande aux collectivités de réduire leurs dépenses, cette hausse de la TGAP va augmenter, inévitablement, le coût du service public de gestion des déchets ménagers, et entraînera donc une augmentation des impôts locaux. Cette hausse sera

la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe des objectifs de développement de la valorisation du biogaz des installations de stockage de déchets non dangereux, la réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement supprime toute incitation fiscale pour ces installations. Elle nuirait ainsi au développement d'une pratique qui permet de réduire le recours aux énergies fossiles, en valorisant l'énergie produite

fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu'elles sont contraintes de traiter des déchets dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. la nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le Gouvernement. Elle pénalisera en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets. Cet amendement vise à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il suit donc le même objectif que les mesures de fiscalité relatives aux déchets proposées par le Gouvernement. Son adoption créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage fixé par le Gouvernement. Cette mesure renforcerait la cohérence du dispositif fiscal présenté par ce dernier : le signal prix sur le stockage, et l'incinération fonctionnerait pour les collectivités qui n'ont pas réalisé les efforts de réduction du stockage,

Il s'agit concrètement d'augmenter progressivement le coût de la mise en place des décharges de déchets, de sorte que celles-ci ne dépassent pas 10 euros la tonne du recyclage. C'est le principe qui était déjà défendu dans les autres amendements. J'ajouterai simplement, et

La réforme proposée supprime progressivement ou diminue fortement toutes les réfactions existant aujourd'hui, alors qu'elles permettent d'encourager des solutions plus vertueuses. J'ai évoqué précédemment les procédures innovantes : je pense que ce sont celles-là qu'il faut soutenir par des mesures fiscales appropriées.

division par deux des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010.

Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l'élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraînera simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets. Cet amendement de bon sens vise donc à prévoir la trajectoire de la TGAP pour les deux ans à venir, afin que l'on puisse mener une réflexion sur les premiers effets de la feuille de route pour une économie circulaire, et donc ajuster la trajectoire de la TGAP. C'est en respectant cette logique que le caractère incitatif de la TGAP sera maintenu.

n° I-55 rectifié. Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de stockage des déchets valorisant 75 % du biogaz. En effet, alors que la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe des objectifs de développement de la valorisation du biogaz des installations de stockage de déchets non dangereux, la réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement supprime toute incitation fiscale pour ces installations. Elle nuirait ainsi au développement d'une pratique qui permet de réduire le recours aux énergies fossiles en valorisant l'énergie produite par les déchets.

à M. Claude Kern. Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative, cette fois-ci pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. L'amendement

fixent à 0,65, et non à 0,7, le seuil de rendement énergétique pour qualifier une « valorisation énergétique élevée ». Dans les faits, cette surtransposition exclurait près des deux tiers des installations concernées et réalisant d'ores et déjà une valorisation énergétique élevée au titre de la législation en vigueur, française comme européenne. C'est pourquoi le présent amendement entend revenir sur cette surtransposition, en prévoyant un seuil de rendement énergétique à 0,65.

vont devoir, dès le 1 janvier 2019, effectuer un mesurage direct des volumes de biogaz captés. Cette obligation, introduite par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2017, entraîne de nouveaux investissements supplémentaires pour les collectivités. Or cette prescription est impossible à mettre en oeuvre dans les délais prévus par la loi. En effet, la plupart des instruments actuellement homologués sur le marché européen ne sont pas adaptés au mesurage du biogaz des installations de stockage, en raison de la composition hétérogène du biogaz et de son caractère Normaliser le matériel disponible sur le marché et en équiper les installations va prendre plusieurs années. Par conséquent, cela signifie que, dès le 1 janvier prochain, la majorité des collectivités propriétaires d'une ISDND, une installation

l'économie circulaire, et donc le recyclage, puis, en deuxième niveau, les unités de valorisation énergétique performantes et, enfin, en troisième niveau, le traitement direct.

Mme Angèle Préville, pour explication de vote. Nous nous devons de ne pas polluer et d'économiser les matériaux, donc de recycler. Or nous continuons à gérer comme avant, et nous faisons face à des problèmes de plus en plus complexes. Nous mettons en place des procédés toujours plus sophistiqués. En vérité, les consommateurs sont captifs et subissent les coûts. Par conséquent, les collectivités sont obligées de gérer des déchets qui leur sont en somme C'est ce qui pose problème. Ce qui serait plus vertueux, plus efficace et permettrait une baisse drastique des déchets serait de prendre le problème véritablement à la racine, c'est-à-dire de limiter en amont les déchets, d'interdire les emballages non valorisables, en plastique notamment, et tous les suremballages, et d'imposer- j'insiste sur ce terme -le compostage des déchets alimentaires, très facile et très peu coûteux à mettre en place. Je

souhaitant bénéficier du taux réduit de TGAP stockage pour la valorisation à 75 % du biogaz capté vont devoir, dès le 1 janvier 2019, effectuer un mesurage direct

Près d'un tiers des déchets ménagers des Français est composé de produits, hors biodéchets, n'ayant pas de filière de recyclage. Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs, la REP. Ils n'ont donc pas d'incitation à se tourner vers l'économie circulaire. C'est une sorte de « prime au cancre la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local. Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euro par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l'amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.

Cet amendement vise à exclure l'huile de palme de la liste des biocarburants éligibles à la minoration du taux de prélèvement supplémentaire à la TGAP, alors que, depuis plusieurs années, son usage comme carburant augmente. Il convient de mettre fin à un signal négatif pour notre environnement en supprimant une niche fiscale dénuée de fondement.

Si l'on prend en compte les changements d'affectation des sols indirects, ou CASI- en d'autres termes, la déforestation -, les biocarburants à base d'huile de palme sont ceux qui ont le pire impact sur le climat. Il s'agit donc d'une différenciation non pas selon l'origine, mais sur le fondement d'un argument environnemental, naturellement compatible avec les règles de D'ailleurs, les États-Unis ont déjà exclu l'huile de palme de leur programme de soutien aux carburants renouvelables, sans pour autant en interdire l'importation. Cet amendement ne tend qu'à anticiper l'application la directive européenne dite RED II, qui prévoit un plafonnement puis une sortie à l'horizon de 2030 des biocarburants à fort risque de La liste de tels biocarburants doit être précisée par un acte délégué de la Commission européenne, en février 2019. Quelle que soit la décision de la Commission, le texte prévoit la possibilité pour les États membres d'aller plus loin dans la différenciation des biocarburants.

Cet amendement vise à insérer un mécanisme de suramortissement de la taxation des hydrofluorocarbures, afin d'aider les entreprises, sans distinction de secteur ni de taille, à investir dans des équipements frigorifiques utilisant des fluides à pouvoir de réchauffement planétaire faible, et donc à moindre impact sur le climat.

a pour objet d'accorder une déduction exceptionnelle, fixée à 40 % de la valeur d'origine des biens- hors frais financiers -acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1 janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, ou commandés

Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation du bien. L'incitation prévue ce suramortissement porte sur l'acquisition à l'état neuf de biens que les entreprises utiliseront durablement dans le cadre de leur activité. Il s'agit donc d'accompagner

C'est un dispositif utile pour les entreprises qui souhaitent s'équiper de technologies alternatives. Avis favorable sur ces deux amendements. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-927

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % aux opérations de prestation de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation-matière des déchets dès 2019, et non à compter de 2021 comme le dispose l'article 59 de ce projet de loi de finances. L'article 8 du texte prévoit une augmentation des taux de la taxe générale sur les activités polluantes due par les installations d'incinération et de stockage à compter de 2021, et une suppression, dès 2019, du taux réduit de TGAP dont bénéficient les installations de stockage répondant à la norme ISO 14001, ce qui conduira à augmenter le taux de TGAP de 33 euros par tonne en 2018 à 41 euros par tonne en 2019 pour environ 20 % de ces installations. Réduire le taux de TVA sur les opérations de tri et de recyclage dès 2019 permettrait par ailleurs de diminuer plus rapidement l'écart de coût entre ces opérations et les solutions de stockage et d'incinération. Tel est l'objet de cet amendement.

pourra être encouragée l'utilisation du compost pour les espaces verts. En ville, le lombricomposteur est une solution au manque de place et est complémentaire aux dispositifs déjà existants dans de nombreuses municipalités de compost collectif. Quel

Nous changeons totalement de sujet ; nous passons des déchets à

présenter l'amendement n° I-600. Je ne reviendrai pas sur les différents éléments que le rapporteur général vient de présenter. Je veux simplement attirer l'attention des membres de notre assemblée

C'est donc à partir d'une analyse technique conjointe que nous convergeons politiquement vers une solution qui doit permettre de faire recouvrer

produisent les recettes que la France est en droit d'attendre. Grâce à ce dispositif, les détenteurs de capitaux qui perçoivent des dividendes et qui trouvent à échapper à la loi fiscale française par des dispositifs éminemment critiquables relevant- cela reste à diagnostiquer -soit de la fraude,

remercier le président de la commission des finances et le rapporteur général d'avoir bien voulu, après de multiples tentatives, créer ce groupe de travail sur la fraude fiscale qui donne aujourd'hui

de finances. Je sais qu'il est un peu tard, mais peut-être M. Darmanin exprimera-t-il son avis favorable par un nouveau tweet, sait-on jamais ? J'espère que nous finirons cette belle soirée en adoptant ce bel amendement.